La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 1 décembre 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. j'ai le profond regret de vous faire part du décès, survenu ce matin, de notre collègue Catherine Fournier, sénatrice du Pas-de-Calais depuis 2017.

Mes chers collègues, par lettre en date du 1 décembre dernier, M. Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste, demande l'inscription à l'ordre du jour de l'espace réservé à son groupe du jeudi 13 janvier de la proposition de loi relative au port du casque à vélo et dans le cadre d'autres moyens de transport, ainsi que de la proposition de loi visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19. Une discussion générale de quarante-cinq minutes est demandée pour chacun de ces textes. Acte est donné de ces demandes. Pour l'examen de ces deux textes, la commission des lois et la commission des affaires sociales se réuniront pour le rapport et le texte mercredi 5 janvier, au matin. Nous pourrions fixer le délai limite de dépôt d'amendements en séance publique au lundi 10 janvier, à douze heures. Il n'y a pas d'opposition ? ... Il en est ainsi décidé. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires Mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'hémicycle, y compris pour les orateurs s'exprimant à la tribune, conformément à la décision de la conférence des présidents réunie le 1 décembre dernier.

car les textes votés par les deux chambres comptaient encore d'importantes divergences. Toutefois, nos échanges fournis, notre travail approfondi, la mobilisation importante de notre commission des affaires économiques et de sa présidente, que je remercie, ont permis de rapprocher progressivement nos positions et, finalement, de trouver un accord, ce dont je me félicite. Cet accord est d'autant plus bienvenu que le texte que nous avons examiné est, nous le savons, très attendu. Nous l'avons constaté lors de nos auditions et nous nous le sommes dit dans cet hémicycle : la régulation du foncier agricole français devait évoluer pour mieux prendre en compte le recours croissant aux sociétés. C'était une nécessité, et le Sénat a soutenu le texte proposé par Jean-Bernard Sempastous, qui visait à apporter une piste de réponse. Dès le début, le Sénat s'est donc inscrit dans une perspective constructive sur ce texte,

Nos deux assemblées ont parfois adopté des approches divergentes, mais nous avons su nous retrouver sur l'essentiel : l'installation des jeunes, la préservation du modèle d'exploitation familiale et la lutte contre la concentration excessive des terres. des terres. C'est là une vraie victoire pour le secteur agricole. Le Sénat a su faire entendre sa voix sur ce texte. Dès l'examen en commission, nous nous étions fixé quatre lignes directrices : territorialiser, recentrer, encadrer et évaluer. Sur chacun de ces points, nous avons réussi à faire évoluer le texte voté par l'Assemblée nationale. J'en citerai quelques exemples. Concernant la territorialisation, nous avons fait « redescendre » la décision, pour que les agriculteurs et les sociétés aient un interlocuteur de terrain ce sera le préfet de département, et non celui de région, qui sera chargé du contrôle sociétaire. Comme nous le souhaitions, le champ du contrôle a été recentré pour viser les transactions excessives et non l'ensemble des cessions. Ainsi, le seuil déclenchant le contrôle a été fixé à 1,5 fois la surface agricole utile régionale moyenne. Nous avons aussi obtenu le maintien des exemptions relatives aux cessions intrafamiliales et conjugales, ainsi qu'entre associés agriculteurs c'était là un apport fondamental du Sénat. Nous avons cependant veillé à bien les encadrer, pour éviter tout contournement. Concernant l'encadrement, nous avons garanti la transparence de la procédure de contrôle et la clarté des rôles de chacun.

Nous avons aussi supprimé l'obligation stricte de passer par la Safer pour réaliser les cessions ou locations prescrites : les parties pourront proposer au préfet des opérations amiables, dès lors qu'elles remplissent le cahier des charges fixé. Nous nous sommes assurés qu'il n'existerait pas de suspicion de conflits d'intérêts à l'égard des Safer, en prévoyant que toute intervention de leur part sur les actifs d'une société dont elles ont instruit le dossier passe par des mesures compensatoires formelles et encadrées, et non par des tractations amiables ouvrant la porte à des dérives. Enfin, la proposition du Sénat de réaliser une évaluation à trois ans de ce nouveau pan de régulation a été unanimement saluée. Elle permettra de dresser un premier bilan et, le cas échéant, d'ajuster les paramètres pour assurer une régulation exigeante, mais équitable. Mes chers collègues, je souhaite le redire devant vous aujourd'hui je suis favorable à une régulation modernisée, complétée, efficace, de l'usage et de la transmission du foncier agricole en France. Cependant cette régulation doit être juste, proportionnée et respectueuse du travail de nos agriculteurs. Elle doit accompagner l'évolution de notre agriculture, mais pas démanteler l'existant ni mettre en danger la viabilité des exploitations. Elle doit être assez souple pour permettre à notre agriculture de s'adapter, tout en étant assez exigeante pour refuser et punir tout abus. Grâce aux nombreux apports du Sénat, le texte de la commission mixte paritaire est équilibré et respectueux des lignes rouges que nous nous étions fixées collectivement. J'adresse une nouvelle fois mes remerciements au rapporteur de l'Assemblée nationale et auteur de la proposition de loi, Jean-Bernard Sempastous, pour nos échanges francs et constructifs qui ont permis d'améliorer le texte. Le travail parlementaire est venu compléter et approfondir l'importante concertation qu'il avait déjà menée ; je pense que nous avons une nouvelle fois démontré toute la pertinence de la navette parlementaire.

de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Je tiens à remercier, à ce titre, le groupe RDPI et son président, François Patriat, d'avoir décidé l'inscription de ce texte dans leur ordre du jour réservé.

Grâce à ces nouvelles dispositions, vous avez fait le choix de renforcer nos outils de politique foncière et de créer un dispositif de contrôle des prises de contrôle des sociétés.

Le premier enjeu était de pouvoir moderniser et adapter nos outils de régulations foncières, afin de garantir dans le long terme l'excellence de la ferme française. Le second enjeu qui nous oblige aujourd'hui est le défi de la transmission.

entre les deux chambres. Le seuil d'agrandissement significatif sera fixé entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne. La pondération, supprimée, aurait suscité une trop grande latitude et une trop grande complexité dans le dispositif, L'exonération familiale a été maintenue au quatrième degré, comme le souhaitait la Haute Assemblée. Pour limiter les effets de cet élargissement, les conditions d'exploitations effectives étaient importantes ; vous avez su les instaurer. prévoir lorsque l'acquisition des titres sociaux est réalisée au profit d'un associé déjà présent dans la société a été maintenue, sous réserve d'une participation effective aux travaux agricoles.

Au regard de ces éléments, je crois que vous avez su trouver, là aussi, un équilibre, qui a d'ailleurs été salué par les organisations professionnelles agricoles. proposition de loi constitue, selon moi, une étape décisive et nécessaire visant à bâtir l'avenir d'une agriculture forte, d'excellence, pourvoyeuse d'emplois pour des femmes et des hommes fiers de leur métier dans nos territoires.

la compétitivité de notre agriculture et l'installation de nos jeunes agriculteurs. Nous passons

et nos déceptions tout au long de l'examen de la proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers des structures sociétaires. Aussi éviterai-je d'entrer trop dans les détails, pour ne rappeler que les faits les plus essentiels et finir par un peu de prospective. Globalement aligné sur la version votée au Sénat, le texte adopté à l'issue du travail conjoint des députés et sénateurs en commission mixte paritaire a permis de faire évoluer certains points : déclenchement du contrôle à 1,5 fois le seuil au lieu de 2 notre groupe souhaitait le déclenchement à 1 fois le seuil ; pas de pondération en fonction du nombre d'associés ; absence de traitement spécifique pour les indivisions ; pas d'exemption pour les salariés d'exploitation agricole en cours d'installation ; pas d'obligation de notification aux interprofessions ; rétablissement, dans une nouvelle écriture, de l'article 5. l'article 5. Quelques-unes des mesures allant dans le sens d'un modèle de ferme que nous connaissons actuellement vers un modèle de type « firme » ont également été maintenues : exemptions pour les cessions intrafamiliales jusqu'au quatrième degré de parenté, ainsi que pour les personnes liées par un possibilité pour les parties de réaliser des compensations amiables sans avis des Safer. Le texte résultant de nos travaux est donc encore plus libéral que celui que nous avons examiné à son arrivée au Sénat. La proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale ne nous convenait pas : elle nous convient encore moins après cette Nous voici encore une fois face à une occasion manquée ! Cette proposition de loi conserve de nombreux angles morts : le détournement du travail à façon et celui du droit des sociétés, deux sujets pourtant cruciaux qui n'ont pas du tout été abordés dans ce texte. Le statut de l'actif agricole, dont nous sommes nombreux à demander la clarification a été, lui aussi, consciencieusement oublié. Deux piliers nous semblent pourtant fondamentaux pour rétablir de l'équité dans la répartition des terres agricoles : le maintien d'une agriculture diverse et familiale au détriment des monopoles et la supériorité du facteur humain face au jeu des capitaux. Sans ces deux conditions, aucune politique des structures responsable ne verra le jour. Et ce n'est certainement pas cette proposition de loi qui nous en donnera l'occasion ! Non, la terre n'est pas une valeur marchande comme les autres. Je rappellerai, sur ce point, la mise en garde d'Edgar Pisani : « Le maintien des biens de la nature parmi les biens marchands nous conduira à l'accélération des phénomènes menaçants dont nous sommes déjà les témoins. » L'accaparement des terres est un phénomène que l'on observe à travers le monde, et bien entendu dans notre pays. Il est le fait non pas seulement de l'avidité d'investisseurs étrangers, aussi de nos propres agriculteurs. C'est une problématique très ancienne, contre laquelle le législateur a toujours lutté. C'est un fait, chers collègues, l'inégalité du partage de la terre et les processus d'accaparement sont des facteurs d'instabilité politique, économique et sociale. L'enrichissement de quelques-uns se traduit par une fragilisation économique collective, et les spécialisations excessives qui en découlent ont des effets négatifs sur le plan agronomique. Dès lors, encourager les dérives du libéralisme en ce qui concerne un bien commun si précieux ne fera qu'accentuer cette instabilité. Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Les Safer ont régulièrement alerté les pouvoirs publics sur les conséquences d'une dérégulation exponentielle, alors que près de la moitié des agriculteurs seront partis à la retraite d'ici à dix ans. Cela ne permettra pas de créer les conditions favorables au développement de l'agroécologie, donc d'obtenir une nourriture de qualité pour tous, tout en protégeant la biodiversité et en luttant contre le changement climatique. Il n'y aura pas d'agroécologie sans relève, et cette dernière sera impossible sans une politique foncière juste. Il faut donc permettre un accès à la terre à la nouvelle génération grâce au partage, au portage et au financement du foncier agricole.

précisé le statut de l'actif agricole et celui du fermage dans sa dimension sociale et environnementale. Par ailleurs, il aurait tendu vers l'objectif de zéro artificialisation nette, avec des règles d'urbanisme cohérentes et une fiscalité limitant la spéculation. moderniser et de démocratiser les instruments de prospective et de mise en oeuvre des politiques foncières. Enfin, parce que nous ne vivons pas sur un continent isolé et que le phénomène d'accaparement des terres, comme je l'ai souligné, se constate dans de nombreux pays, parfois à des degrés encore plus inquiétants qu'en France, un tel texte aurait mis l'accent Cette idée rejoint un principe simple qui devrait d'ailleurs figurer dans la loi : le sol, comme les autres ressources naturelles, est un bien qui ne saurait profiter à quelques-uns au détriment de tous. Tel est le voeu de nombreuses organisations professionnelles, des représentants des collectivités territoriales et des ONG, mais aussi d'une part de plus en plus grande de nos concitoyens. C'est aussi le nôtre. et Républicain persistera donc à désavouer ce texte qui ne correspond en rien aux principes je viens d'énoncer, lesquels nous paraissent pourtant fondamentaux pour répondre aux enjeux de notre agriculture et préserver nos terres agricoles. Mes chers

Que de succès, mes chers collègues !

Notre rapporteur, Olivier Rietmann, a été lui aussi maître dans l'art de la négociation. Il a su convaincre le rapporteur de l'Assemblée nationale des apports du Sénat, qui ont souvent été compris par la majorité au Palais-Bourbon. Jean-Bernard Sempastous et Nicolas Turquois, constructifs et pragmatiques dans leur approche, n'ont pas démérité et ont su avancer sur toutes les lignes qui paraissaient encore difficilement franchissables

Chacun a su faire un pas vers l'autre, ce qui nous a permis, finalement, de parvenir à un texte une nouvelle fois salué par les organisations interprofessionnelles concernées. Parmi les principaux compromis à souligner, je reviendrai sur le seuil de déclenchement grâce auquel le préfet actera le contrôle des cessions de parts sociétaires.

Concernant les exemptions, c'est le Sénat qui a été écouté. Elles s'étendent jusqu'au quatrième degré, pour y inclure les cessions aux cousins germains. De même, nous accordons ce bénéfice aux couples mariés et pacsés, ainsi qu'aux associés dès lors que ceux-ci sont exploitants à titre principal. Pour ce qui est du dispositif des mesures compensatoires, la compensation pourra naturellement passer par la Safer, mais elle pourra aussi avoir lieu par voie amiable avec le préfet, si le demandeur souhaite la réaliser seul en proposant un candidat. un candidat. Les députés ont souhaité qu'une attestation de réalisation des engagements soit apportée par le pétitionnaire pour que la cession de part soit bien valide. compromis sur le point le plus ardu des discussions, à savoir la non-intervention commerciale des Safer sur les dossiers qu'elles ont instruits. Là encore, chaque partie a su faire preuve d'une grande sagesse. grande sagesse. L'impossibilité faite aux Safer d'intervenir sur les dossiers sera limitée à un an, au lieu des neuf années initialement prévues ; un certain nombre de dérogations à cette règle laissent penser que le sujet est suffisamment encadré. Enfin, à la demande de la majorité de l'Assemblée nationale, l'article 5 a bien été rétabli, mais remanié. Le dispositif vise à renforcer l'efficacité du contrôle des structures, en permettant au préfet de renforcer ses prérogatives.

Ce délai allongé permettra de laisser plus de temps à d'autres candidats pour se positionner. Ces compromis nous semblent justes, pertinents et équilibrés. En définitive, le texte de Jean-Bernard Sempastous, qui porte cette réforme depuis de longues années, est une étape décisive pour l'accès au foncier agricole, en direction de nos jeunes agriculteurs. Ne boudons pas ce plaisir et félicitons-nous de ce travail transpartisan ! Continuons sur ce chemin vertueux en vue du projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Bien évidemment, notre groupe votera le texte issu des

Le foncier agricole est un sujet urgent sur l'ensemble de notre territoire. Il l'est à plusieurs niveaux. Face à l'artificialisation grandissante des sols dans notre pays et à l'évolution des formes d'exploitation, nous devons préserver ce foncier agricole pour notre souveraineté alimentaire actuelle, mais surtout pour celles des générations futures. En Haute-Garonne, notre activité agricole est un moteur de vie et d'entretien des espaces naturels. Plus de la moitié de la surface de mon département est cultivée ou en herbage pour l'élevage. Cela concourt à maintenir notre souveraineté alimentaire, notre culture gastronomique incomparable et nos emplois sur un territoire fragilisé. Nous sommes fiers de nos agriculteurs et de leur savoir-faire. Nous sommes également fiers des évolutions positives qu'ils font vivre aux systèmes agricoles. Très tôt, l'enjeu du foncier a été posé en France. Nous avons construit des outils de régulation, cités en exemple par nombre d'autres pays. Force est de constater que ces outils, bien qu'ils soient efficaces, doivent être adaptés aux évolutions actuelles. Notre groupe demeure favorable à une solution d'équilibre entre la nécessaire liberté d'entreprendre et la sécurité issue d'une régulation ajustée.

Nous trouvons aujourd'hui des solutions pour le foncier agricole, mais demain des dossiers tels que le statut de l'exploitant ? Nous appelons donc encore de nos voeux une grande loi agricole et nous resterons attentifs à la suite qui sera donnée à ces dossiers.

Il est particulièrement nécessaire en ce qu'il permettra une véritable évaluation des dispositions mises en place. Il comportera également de potentielles recommandations sur les évolutions à mettre en oeuvre. Les enjeux liés à l'installation des jeunes et à la transmission familiale des exploitations connaissent également des avancées intéressantes. Je salue la préservation du quatrième degré concernant l'exonération au dispositif de contrôle des cessions de parts sociétaires que met en place cette

Les réalités du monde agricole n'ont jamais été aussi visibles : la place cruciale qu'il occupe a été particulièrement mise en lumière par la crise que nous vivons. La protection de notre foncier agricole participe à la préservation de notre souveraineté alimentaire et de notre tradition agricole française.

Gardons en tête qu'il ne représente que l'une des premières étapes d'un long travail à poursuivre. Soyez certains que nous serons au rendez-vous ! La parole

sûr ! ... permet de rapprocher la décision du territoire, de garantir la fluidité des transactions tout en les contrôlant pour garantir un meilleur fonctionnement du marché foncier agricole

monsieur le ministre, mes chers collègues, comme en première lecture, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne peut que faire part de sa déception sur la proposition de loi, qui ne parviendra pas à mettre en place une régulation efficace et équitable de l'accès au foncier, pourtant nécessaire à la transition de notre système agricole. Un accès partagé aux terres agricoles est en effet un enjeu majeur à l'heure du renouvellement des générations et du développement d'une financiarisation du foncier qui menace l'installation et la consolidation de fermes familiales, à taille humaine. Certes, cette proposition de loi vient répondre à une véritable problématique : l'absence de contrôle sur les transferts de parts de sociétés agricoles, qui permettait de contourner les dispositifs de régulation que sont la Safer et le contrôle des structures, ouvrant ainsi la voie à une concentration foncière importante. pour corriger cet angle mort de la réglementation, la voie choisie dans ce texte est l'instauration d'un dispositif de contrôle faible, incomplet et trop facilement contournable, qui sera donc au mieux inefficace, au pire contre-productif. En effet, notre diagnostic reste le même qu'en première lecture : l'institutionnalisation d'un système de deux poids deux mesures entre le contrôle s'appliquant aux sociétés et celui des personnes physiques, c'est tout le système de régulation foncière qui est affaibli. nous, le seuil de déclenchement du contrôle devrait être identique à celui du contrôle des structures, à la fois pour garantir une égalité de traitement et pour proposer une véritable régulation.

commission mixte paritaire conserve de nombreuses exemptions permettant d'échapper au contrôle, dont une partie, ajoutée par le Sénat, autorisera des agrandissements, notamment au moment du départ à la retraite d'associés. De plus, le système de mesures compensatoires qui est proposé reste pour nous inacceptable. Sur le principe, nous n'étions pas d'accord avec l'idée de donner un blanc-seing à de grands agrandissements, sous prétexte de laisser quelques hectares pour une installation.

Avec ce texte, je crains que les garde-fous ne soient insuffisants pour éviter ces dérives. Enfin, la rédaction de l'article 5 est pour nous un recul par rapport à sa version initiale : un délai supplémentaire pourrait ne pas suffire à débloquer des situations où ce sont des prix dissuasifs qui découragent les candidatures concurrentes. Cette mesure peut constituer une modeste amélioration, mais nous regrettons que la version de l'Assemblée nationale, seule véritable avancée du texte pour l'installation, n'ait pas été conservée. Par ailleurs, comme nous l'avions souligné en première lecture, le fait que le texte ne comporte pas de dispositions sur le travail délégué ou sur les investissements étrangers contribue, là aussi, à lui faire rater sa cible. cible. Nous partageons le constat d'organisations agricoles et d'ONG, qui estiment que le texte ne permettra pas de renverser la tendance à l'agrandissement des fermes, tendance qui, malheureusement, continuera également d'être nourrie par la nouvelle PAC, avec les conséquences que l'on connaît pour l'emploi paysan et la vie des territoires. Alors que les consommateurs réclament des productions locales diversifiées et de qualité, ainsi que des paysages préservés et riches en biodiversité, et alors que de plus en plus de porteurs de projet, souvent non issus du milieu agricole, souhaitent répondre à cette demande, nombre d'entre eux renonceront à leur projet faute de trouver des terres pour s'installer. C'est toute une dynamique présente sur les territoires qui ne demande qu'à être encouragée, et que ce texte ne viendra pas accompagner.

une politique qui permette d'assurer, par la multiplication de fermes diversifiées et à taille humaine, notre souveraineté alimentaire et la transition agroécologique. Ce texte constitue, à cet égard, pour reprendre les mots de notre collègue Christian Redon-Sarrazy, une occasion manquée, et c'est donc avec regret que nous nous y opposerons une nouvelle fois.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous l'avions dit lors de l'examen de cette proposition de loi, si nous avons conscience

Ainsi, comme de nombreux observateurs, nous pensons que le remède pourrait être pire que le mal, puisque nous créons finalement un système de deux poids deux mesures, en lieu et place d'un même seuil de contrôle pour tous et d'arbitrages reposant sur un corpus législatif commun. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi est opérée une distinction entre le seuil général de contrôle des structures et le seuil qui qui s'appliquera aux sociétés, ni pourquoi il a été choisi de mettre en place une inégalité de traitement entre les personnes physiques et les personnes morales détentrices de parts de sociétés. Cela risque d'accélérer le phénomène sociétaire, donc, inévitablement, l'agrandissement que cette proposition de loi est pourtant censée combattre. Pis, ce texte instaure de multiples dérogations au nouveau contrôle des cessions des parts sociales, voire un cumul des différentes dérogations permettant l'agrandissement sans contrôle d'une exploitation. Lors des débats en première lecture, il avait été rappelé, à juste titre, qu'« il suffirait de se pacser avec son salarié qui est aussi son cousin éloigné Sans parler de la mise en place de mesures compensatoires qui permettront l'agrandissement, mais aussi l'accélération de la financiarisation de notre agriculture et mettront à mal les contrôles traditionnels faut-il se contenter d'une loi sur le foncier, au risque de ne plus aborder ce sujet pourtant fondamental ? Faut-il se contenter d'un compromis qui, malheureusement, n'endiguera pas le phénomène de libéralisation qui ne garantira pas un accès et un usage équitables à ce bien commun, même si certains n'aiment pas cette expression, qu'est le foncier agricole

Terres de Liens, la Fédération nationale d'agriculture biologique, aGter et France Nature Environnement, tous dénoncent le manque d'ambition du texte, qui « ne réglera aucunement la difficulté d'accès au foncier [ ...] pour les porteuses et porteurs de projets agricoles et notamment les " non-issus du milieu agricole " ». Or, comme le soulignent un certain nombre de spécialistes du droit du foncier agricole, le foncier constitue la trame essentielle du territoire que le code de l'urbanisme qualifie de « patrimoine commun de la Nation ». Et, ne nous y trompons pas, sur ce sujet comme sur bien d'autres, nombreux sont ceux qui plaident pour la disparition de toute régulation au motif qu'elle serait un frein à la liberté d'entreprendre et au développement économique des entreprises agricoles, tout cela au nom de la compétitivité. En

l'agrandissement excessif des structures, la diminution du nombre d'exploitations et d'exploitants et l'industrialisation des processus de production ont des conséquences néfastes pour l'aménagement du territoire, l'environnement, la qualité des produits et des sols, l'emploi et, surtout, la vitalité des territoires ruraux. L'accaparement des ressources foncières, par des investisseurs étrangers, mais aussi par de grands groupes nationaux, nationaux, représente une véritable menace. Nous pouvons toutes et tous, en tant que de besoin, le dénoncer. Malgré ce constat, permettez-moi permettez-moi de le dire, nous restons en deçà des enjeux, nous nous éloignons toujours plus du « pacte foncier qui, depuis les années 1960, établit dans le monde agricole un équilibre entre la propriété

les Jeunes Agriculteurs se sont mobilisés pour distribuer gratuitement aux passants plus de 1 100 baguettes de pain, correspondant à la production perdue toutes les minutes du fait de la disparition de foncier agricole- un symbole très fort, vous en conviendrez Cette opération avait pour objectif de faire « prendre conscience aux consommateurs que si, demain, il n'y a plus de foncier agricole, il n'y aura plus de production alimentaire en France ». Le Sénat salue l'initiative de cette proposition de loi, qui atténuera la disparition du foncier. Il s'agit ici de relever le défi de la maîtrise du foncier aux moyens de deux objectifs lutter contre la concentration excessive des exploitations et l'accaparement des terres, en contrôlant les cessions de titres des sociétés ; d'autre part, agir pour l'installation et la consolidation des exploitations, grâce à un mécanisme d'incitation à vendre ou à donner à bail rural à long terme une surface compensatoire à un agriculteur. Le coeur du dispositif, créé à l'article 1, est inspiré de celui de l'Autorité de la concurrence pour le contrôle des concentrations économiques. Il instaure un contrôle administratif et des prises de participations sociétaires, au profit d'un bénéficiaire qui dépasse un seuil d'agrandissement significatif. mercredi 1 décembre, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord après des heures de négociation déterminées et des prises de position solides. Elle a conforté les mesures votées par le Sénat en novembre. Nous avons maintenu Nous avons maintenu l'essentiel de nos positions d'équilibre visant à réguler sans faire obstacle au développement de notre secteur agricole. Ainsi, le préfet de département sera compétent pour conduire la procédure de contrôle, au plus près des exploitants et de leur activité, reprenant ainsi une proposition du Sénat. Le préfet de région est toujours chargé de fixer le niveau du seuil. Le seuil plancher déclenchant le contrôle des cessions a été rehaussé à 1,5 fois la surface agricole utile régionale moyenne, conformément à la volonté du Sénat de viser les opérations excessives, et non la majorité des opérations courantes. Les transmissions entre membres d'une même famille, dès lors qu'ils s'engagent à poursuivre l'exploitation, ont été exclues du dispositif de contrôle jusqu'au quatrième degré inclus, comme l'avait prévu le Sénat. Pour ne pas complexifier à outrance le travail des agriculteurs qui ont choisi de s'associer au sein d'une même société, les transmissions entre exploitants associés de longue date ont été permises, mais encadrées. L'accord qui a été trouvé reconnaît la liberté de gestion des agriculteurs dans la mise en oeuvre des mesures compensatoires, en leur laissant la possibilité de proposer au préfet un locataire ou un acheteur pertinent, ou d'opter pour l'appui de la Safer. De manière unanime, les membres de la commission mixte paritaire ont soutenu la volonté du Sénat de demander au Gouvernement une évaluation obligatoire, précise et chiffrée de ce nouveau dispositif de contrôle d'ici à trois ans. L'article 5, qui vise le cas d'un acquéreur unique, a été rétabli par la

Afin de rendre opérationnelles ces mesures d'urgence au plus vite, la commission mixte paritaire a prévu une entrée en vigueur de l'article 1 à une date fixée par décret, au plus tard le 1 juillet 2022. Les agriculteurs attendaient une grande loi. Ce n'est pas le grand soir du foncier agricole, chacun en convient ! Même si les débats ont été vifs entre les deux chambres, même si des discordances ont pu se faire entendre parmi les acteurs de la filière,

En effet, si nous voulons avoir un minimum de souveraineté alimentaire, si nous voulons une agriculture durable, diversifiée et des produits de qualité, si nous voulons sécuriser l'emploi agricole et garantir ainsi le dynamisme de nos territoires ruraux, nous sommes bien d'accord il faut absolument préserver un modèle équilibré, dans lequel coexistent des exploitations de taille différente, des exploitations sous forme sociétaire et surtout des structures familiales, qui, au-delà d'une communauté de travail, représentent bien souvent une communauté de vie. de vie. À l'issue de l'examen de la proposition de loi de notre collègue député Jean-Bernard Sempastous, nous allons, je le crois, dans le sens de cet objectif, même si les défis de la politique foncière appellent une réflexion plus vaste que le seul contrôle des structures et cessions de titres sociaux.

réformer. En attendant, nous avons aujourd'hui la possibilité d'apporter un début de réponse à une évolution observée dans nos régions, celle de la part de plus en plus importante des formes sociétaires au sein de notre modèle agricole. On en connaît les conséquences : l'accaparement des terres et les difficultés d'accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, alors même que près d'un agriculteur sur deux atteindra l'âge de la retraite au cours des cinq à sept prochaines années, comme cela a été souvent rappelé dans nos débats. La Safer, compétente en la matière, doit pleinement faire de l'installation sa priorité. Monsieur le ministre, il faudra pour cela lui donner les moyens nécessaires. L'adaptation rapide du contrôle des cessions de parts de sociétés s'impose donc. Aussi, mon groupe partage tout à fait l'ambition de cette proposition de loi. Je suis heureux de constater que la commission mixte paritaire a trouvé un équilibre satisfaisant, préservant au passage les quelques apports du RDSE. Je ne reviendrai pas sur la question du seuil surfacique, qui a été très discutée. Je rappellerai seulement que j'aurais préféré que l'on s'en tienne à la fourchette fixée dans le texte initial, un niveau qui me semblait bien répondre à la diversité des exploitations couvrant notre territoire. J'approuve également l'encadrement des exemptions au contrôle. Je note toutefois que celles-ci demeurent nombreuses, et qu'un effort n'a pas été fait en direction des foncières agricoles agréées entreprises solidaires d'utilité sociale ». Nous sommes quelques-uns ici, y compris le Gouvernement, à avoir souligné notre attachement à Terre de Liens, qui effectue un travail remarquable de promotion des exploitations durables et sociales. Enfin, la clarification de la procédure pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires, ainsi que le rétablissement sur la base d'une nouvelle rédaction de l'article 5, relatif à l'adaptation des motifs de refus d'autorisation d'exploiter, permettent de retrouver l'esprit de la proposition de loi initiale. Mes chers collègues, compte tenu des améliorations apportées par la commission mixte paritaire, le RDSE approuvera ce texte. Sans anticiper les prochains débats, je me réjouis également de l'examen après-demain de la proposition de loi sur les retraites agricoles, puis à la rentrée du grand projet de loi sur l'assurance récolte. Protéger le foncier agricole, protéger les agriculteurs, qu'ils soient anciens ou actifs, tout cela participe d'une même ambition, celle de conserver à notre pays sa vocation de nation agricole. Conformément

Cette commission mixte paritaire m'a appris une chose dont j'étais convaincu : il ne faut jamais lâcher, surtout dans la dernière ligne droite.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,

les « thérapies de conversion » constituent des atteintes insupportables à l'intégrité humaine. Elles sont totalement inacceptables en France en 2021. Être une personne LGBT+ n'est pas une idéologie. Être soi n'est pas un crime. Non, l'homosexualité et la transidentité ne sont pas des maladies que l'on pourrait soigner. Non, il n'y a rien à guérir, parce que l'on ne choisit pas son orientation sexuelle et parce que l'identité de genre n'est ni plus ni moins que l'identité que l'on ressent au fond de soi. Ces pratiques rétrogrades appelées « thérapies de conversion » embrassent un large spectre de pratiques et revêtent un caractère protéiforme : harcèlements, agressions physiques, exorcismes, retraites spirituelles, traitements hormonaux, et même, parfois, électrochocs. Faire subir des électrochocs à des personnes souvent vulnérables, avec l'illusion de pouvoir transformer ces personnes en ce qu'elles ne sont pas comment l'accepter ? Comment ne pas voir cette vulnérabilité qui se mue parfois en culpabilité, toujours dans une souffrance extrême ? Grâce au travail mené par Laurence Vanceunebrock, en étroite concertation avec des associations, des experts, des médecins et des autorités religieuses, cette proposition de loi instaure un délit spécifique visant à réprimer ces pratiques. L'objectif est de mieux identifier ce délit, de mieux protéger les victimes, de favoriser la libération de la parole et, ainsi, de mieux mesurer l'ampleur de ce phénomène dans notre pays. Oui, cette proposition de loi permettra aux victimes de passer plus facilement la porte des commissariats ou des gendarmeries. Elle permettra aux forces de l'ordre et aux magistrats de mieux appréhender les fautifs, pour mieux les condamner. Ces pratiques ne sont pas nouvelles et dépassent nos frontières. D'autres pays européens, tels que l'Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas, ont déjà légiféré ou sont en train de le faire. Cette loi permettra enfin d'envoyer un signal clair à celles et à ceux qui cherchent à contraindre une personne à renier son identité de genre ou son orientation sexuelle. Cette loi permettra d'envoyer un signal fort aux victimes de ces pratiques, qui, à l'heure actuelle, n'ont pas pas toujours conscience de l'illégalité de ces actes. Par cette loi, nous leur affirmons clairement qu'elles seront protégées. Mesdames, messieurs les sénateurs et les sénatrices, il est important de préciser que les « thérapies de conversion qu'elles soient religieuses, médicales ou sociétales, sont le fait d'une minorité de personnes. Mais cela n'atténue en rien leur gravité. Cette proposition de loi ne vise évidemment pas à stigmatiser celles et ceux qui accompagnent de manière bienveillante les personnes qui en manifestent la volonté. Les aides apportées par la famille ou les amis, le travail accompli par les médecins, les représentants de culte ou les associations restent essentiels et doivent perdurer. L'accompagnement offert à une personne en réflexion sur son orientation sexuelle ou son identité de genre n'est clairement pas visé par ce texte. Notre démarche vise en revanche à renforcer les droits et la protection des personnes LGBT+. L'écoute, le soutien et la protection, d'où qu'ils viennent, sont indispensables. Au moment où les droits des personnes LGBT+ sont remis en cause au sein même de l'Europe, que ces enjeux affleurent dans notre débat public, ce texte s'inscrit dans le combat mené depuis le début de notre mandat contre toutes les formes de discriminations et pour l'égalité des droits de tous les citoyens. Cela se traduit dans le plan triennal d'actions du Gouvernement pour l'égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ lancé le 14 octobre 2020. Ce progrès s'est également traduit par l'ouverture de la PMA (procréation médicalement assistée) aux couples de femmes et aux femmes célibataires, par la publication il y a quelques mois d'une circulaire du ministère de l'éducation nationale pour mieux accueillir les élèves transgenres, mieux appréhender la transidentité et, ainsi, lutter contre le taux de suicide quatre à sept fois plus important pour les personnes concernées. Il se traduit par le renforcement de la formation tant des forces de l'ordre que de la magistrature, par la désignation de référents discriminations au sein du ministère des armées, ou encore par le lancement d'une campagne de communication nationale de lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre par Santé publique France.

Mesdames, messieurs les sénateurs et les sénatrices, il est du devoir de l'exécutif comme du législateur de protéger toujours plus nos concitoyens. Il est du devoir des responsables politiques de prendre en considération

Je voudrais également, devant vous, remercier l'ensemble des associations qui oeuvrent chaque jour pour faire avancer les droits des personnes LGBT+, en particulier celles qui se sont engagées depuis plusieurs années dans ce combat contre les « thérapies de conversion ». Je pense notamment au collectif « Rien à guérir dont le porte-parole Benoît Berthe est présent au Sénat cette après-midi. Monsieur Berthe, je sais le travail que vous avez mené et les obstacles auxquels vous avez été confrontés. Votre contribution est précieuse pour toutes les victimes. Il s'agit pour elles d'une grande avancée. Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs et les sénatrices, je vous remercie toutes et tous pour votre implication et votre travail sur ce texte, en particulier vous, madame la rapporteure Dominique Vérien.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, j'ai une confidence à vous faire en tant que parlementaire, il m'arrive parfois de ne pas saisir pleinement l'intérêt de certains textes, tant ce que l'on veut nous faire voter est déjà présent d'une façon ou d'une autre dans nos codes. À quoi bon créer un nouveau délit alors que les faits sont déjà sanctionnables sur le fondement de dispositions déjà existantes ? ce raisonnement au texte que nous examinons aujourd'hui. On pourrait facilement le balayer et le rejeter d'emblée, en estimant que, de toute façon, les « thérapies de conversion » peuvent d'ores et déjà être sanctionnées par les articles du code pénal relatifs aux violences volontaires, au délit d'abus de faiblesse, au harcèlement moral ou encore à l'exercice illégal de la médecine. Pourtant, il n'en est rien, parce que le droit et la loi ne sont pas des sciences froides et purement objectives. Ils sont aussi le reflet d'une société, de son état d'esprit, de ses valeurs, des interdits qu'elle pose et des choses qu'elle nomme. Car tout l'enjeu de ce texte est bien là et tient en un seul mot : nommer. Nommer le délit, c'est poser une interdiction franche et c'est reconnaître le mal qui a été fait. Nommer le délit, c'est permettre aux victimes de se reconnaître en tant que telles- on sait l'importance que cela peut avoir dans leur reconstruction. Nommer le délit, c'est enfin permettre une véritable quantification du phénomène et une meilleure prise en charge judiciaire. Finalement, c'est un message fort que la République envoie en créant un délit autonome visant à sanctionner les thérapies de conversion. Ces actes ne sont plus acceptables. Peu importe son orientation sexuelle ou son identité de genre, chacun a le droit à la protection de la République. Accepter l'autre au-delà de ses différences, c'est aussi contribuer à faire de notre société un espace de liberté. Ce texte est donc nécessaire. De plus, il s'inscrit dans la continuité de la résolution du Parlement européen du 1 mars 2018 condamnant les thérapies de conversion et appelant les États membres de l'Union européenne à légiférer pour les interdire.

Je voudrais également préciser qu'il ne s'agit pas d'un texte sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Je connais les doutes de certains d'entre vous sur cette dernière qui figure pourtant déjà dans le code pénal, dans le code du travail ou encore dans le code du sport. En outre, le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2017, a estimé que l'expression « identité de genre » était suffisamment claire et précise pour figurer dans la loi. J'ajoute également que les responsables des cultes que nous avons auditionnés et auxquels nous avons clairement posé la question nous ont expliqué non seulement être pour cette loi, mais aussi ne pas avoir de problème avec la présence de la notion d'identité de genre dans le texte. Enfin, le médecin spécialiste que nous avons auditionné a insisté sur le fait que cette réassignation est, dans certains cas, un besoin vital, une question de survie même. ici, la présence de l'expression « identité de genre » sert simplement à protéger ceux qui en ont besoin de ceux qui considèrent qu'homosexualité et transidentité sont des maladies ou des péchés que l'on peut traiter par de pseudosciences. Concrètement, on parle ici de pratiques pouvant prendre la forme de groupes de parole où l'on doit se mettre à nu, de jeûnes, de sessions d'enseignement, de prières de guérison ou de délivrance, d'hypnose, d'électrochocs, voire d'exorcismes, de « viols de guérison »- curieux concept -, ou d'excision. Sauf que, en réalité, il n'y a pas davantage de malades que de maladies. Il n'y a donc rien à guérir. Les seules thérapies possibles sont celles qui visent à soigner les conséquences de ces pratiques barbares et moyenâgeuses. Isolement, dépression, suicide, voilà les seuls résultats que peuvent espérer obtenir ces charlatans. Le constat est dur, mais il est partagé par les associations de victimes bien sûr, mais aussi par les responsables des cultes, qui ont tous tenu à dénoncer les thérapies de conversion, ne serait-ce que parce que ces dernières passent par des dérives sectaires et un profond dévoiement des textes sacrés. Tous ont tenu également à saluer la nécessité Les médecins et les psychiatres nous ont, pour leur part, alertés sur les conséquences désastreuses de ces pseudo-thérapies- je les ai déjà évoquées -, comme sur la nécessité d'offrir une écoute attentive et bienveillante face aux questionnements sur son orientation sexuelle ou son identité de genre. Une écoute bienveillante et attentive est nécessaire, et nous avons justement tenu à rassurer en inscrivant dans ce texte une distinction entre les « thérapies de conversion », que nous condamnons, et l'accompagnement et le soutien. ou le professionnel de santé qui invite à la prudence et à la réflexion le mineur qui s'interroge sur son identité de genre et envisage un parcours médical ne pourra évidemment pas être poursuivi. ne s'agit pas de pénaliser celui qui invite simplement à prendre le temps de la réflexion avant de se lancer dans un changement profond. Il ne s'agit pas non plus ici de pénaliser l'accompagnement spirituel et religieux. La liberté de culte est parfaitement respectée respectée et préservée. Cet accompagnement, qu'il vienne d'un parent, d'un médecin ou d'un proche de confiance, est donc parfaitement légitime, mais il ne doit jamais aboutir à la proposition d'une thérapie de conversion, d'une pratique ayant pour effet une altération de la santé physique ou mentale de la personne. D'ailleurs, dans le cas où cette pratique serait à l'initiative du parent, le juge devra se prononcer systématiquement sur le retrait ou non de l'autorité parentale. Nous estimons qu'il s'agit d'une mesure de bon sens, qui permet d'avoir un texte équilibré et qui s'inscrit dans la continuité du travail de l'auteure de la proposition de loi, Laurence Vanceunebrock, dont je salue ici l'engagement sur le sujet. En définitive, je l'ai dit, ce texte est nécessaire. Alors que ces thérapies de conversion visent principalement des adolescents et de jeunes adultes, à une période de leur vie pleine de questionnements et de doutes, où ils sont bien souvent vulnérables, la République se doit de les protéger. Nous leur devons la possibilité de s'épanouir librement et de se construire. Je m'adresse à tous ceux qui ont été victimes, à tous ceux qui ont eu le courage de témoigner, comme aux anonymes : nous reconnaissons votre peine et nous sommes aujourd'hui pleinement à vos côtés.

le rappeler ? Ensuite, ces réalités renvoient à l'intime de chaque vie. Enfin, au-delà de la dimension politique faisant écho à la mobilisation d'un collectif du même nom, ces trois mots revêtent le caractère de l'évidence, car ils traduisent la réalité des textes français et internationaux. L'OMS a rayé depuis quelques années l'homosexualité et la transidentité de la liste des maladies mentales. Plus encore, l'homophobie et la transphobie sont désormais pénalisées pour ce qu'elles sont : des atteintes au respect et à la dignité de la personne humaine auxquelles notre état de droit ne peut consentir.

Ce texte a ainsi pour objectif que l'application du droit pénal à ces pratiques barbares ne souffre d'aucune de ces ambiguïtés en conséquence desquelles de trop nombreux cas ont été ignorés ou mal appréhendés, parfois même par les victimes elles-mêmes. La proposition de loi s'attaque donc clairement à ces thérapies de conversion, qu'elles se présentent sous une forme religieuse, médicale ou sociétale, en créant deux nouvelles infractions qui posent un interdit explicite assorti de sanctions importantes et aggravées, notamment lorsque la victime chers collèges, ce texte est l'aboutissement d'un travail de conviction de notre collègue députée Laurence Vanceunebrock, qui a été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale ; ce point est suffisamment rare pour être souligné et salué.

Les travaux de qualité de notre rapporteure Dominique Vérien s'inscrivent dans une démarche constructive autour du constat partagé de la nécessité d'agir. Ce texte permettra d'affirmer un interdit fort et d'assurer une meilleure protection et une meilleure prise en charge des victimes. Il permettra également de mieux connaître et quantifier ces pratiques inacceptables pour notre société, afin d'y apporter une réponse adaptée.

Ce texte n'a pas non plus d'incidence sur les pratiques médicales tendant au changement de sexe, comme cela a bien été rappelé à l'Assemblée nationale. Il nous semble à ce titre que des précisions que des précisions sur le champ d'application de la proposition de loi, dans un sens comme dans l'autre, risqueraient de nuire à la clarté et à la bonne application du dispositif adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, mais nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen des amendements. Notre rapporteure a par ailleurs fait oeuvre utile en réinsérant des dispositifs sur le retrait de l'autorité parentale ou en introduisant à l'article 3 des circonstances aggravantes lorsque les thérapies de conversion sont conduites par des professionnels de santé

La transidentité existe dans la réalité des vies et de notre société. Plus encore, elle fait l'objet de ces thérapies de conversion que nous sommes tous résolus à combattre par la loi. L'identité de genre est enfin déjà présente dans le code pénal pour définir les discriminations. Gisèle Halimi disait que « la norme sexuelle ne se définit pas ». Notre objectif de législateur n'est pas ici de la définir. Le sujet ne relève pas de la terminologie : ne nous trompons pas de débat. La proposition de loi que nous examinons cette après-midi est un texte de dignité, juste et ambitieux pour la protection de toutes les victimes de toutes les formes de thérapies de conversion.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, partisans de la démocratie libérale, nous croyons que les libertés individuelles sont essentielles à notre société. Nous croyons que les minorités doivent être protégées. Or la plus petite des minorités, c'est l'individu. Il doit être protégé contre les ingérences d'autres membres de la société dans ce qui relève de sa sphère individuelle. Nous croyons au libre arbitre et nous pensons qu'il y a des décisions que seul l'individu a la légitimité de prendre, qu'il y a des sujets sur lesquels il a seul le pouvoir de se prononcer. Tel est évidemment le cas de la décision du changement de sexe ou du sujet de l'orientation sexuelle. Il faut rappeler que, pendant très longtemps et jusqu'à récemment, ce n'était pas le cas. Nous avons tous en tête le fait que, dans notre pays, l'abrogation des dispositions pénales incriminant les actes homosexuels entre adultes consentants ne date que de 1982. L'homosexualité a officiellement cessé d'être classée comme une maladie mentale il y a une quarantaine d'années seulement. Il est temps que chacun reconnaisse que l'orientation sexuelle d'un individu ne concerne que ledit individu, de même que son identité de genre. Nous croyons aussi que seul cet individu peut légitimement prendre la décision d'un changement de sexe, en conscience et sans contrainte.

Nous nous félicitons de l'initiative prise par nos collègues députés. Nous saluons le travail de la rapporteure sur ce texte et soutenons très majoritairement la position de la commission. Nous sommes sensibles au fait que la rapporteure ait souhaité distinguer clairement les conseils donnés à une personne qui s'interroge sur un éventuel changement de sexe des actes qui portent atteinte à la santé de la victime. Cette précision nous semble tout à fait opportune : les conseils appelant une jeune personne désireuse de changer de sexe à la prudence et à la réflexion ne doivent pas être constitutifs, en eux-mêmes, d'une infraction. Les parents sont toujours attentifs à l'évolution de leur enfant, en particulier dans la phase délicate de l'adolescence. Cependant, lorsque le parent inflige à son enfant une thérapie de conversion qui porte atteinte à sa santé, la question du maintien de l'autorité parentale se pose. Le juge doit pouvoir décider en fonction des conditions de l'espèce si un retrait se justifie.

le texte qui nous est proposé aujourd'hui, en procédure accélérée, affirme la nécessité de lutter contre la non-acceptation de l'homosexualité dans la société, ce qui est effectivement indispensable. Plus précisément, cette proposition de loi tend à interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle. On ne peut en effet ignorer la détresse des hommes et des femmes dont l'orientation sexuelle n'est pas acceptée. Nous leur devons écoute et soutien. Il est essentiel de défendre le droit à la différence et de protéger toutes les personnes injustement traitées, dont certaines sont contraintes de subir ces pratiques. Non, l'homosexualité et la transidentité ne sont pas des maladies à soigner. Nous devons lutter contre toute dérive religieuse, sectaire, familiale ou autre visant à faire croire aux jeunes et aux adultes qu'ils sont malades parce qu'ils ont d'autres orientations sexuelles. sexuelles. Plusieurs pays ont légiféré récemment en matière de thérapies de conversion. La chambre basse canadienne vient ainsi de voter une loi interdisant les thérapies de conversion. De même, les thérapies de conversion pour personnes homosexuelles vont être interdites en Angleterre et au Pays de Galles. Galles. Si la notion d'orientation sexuelle est claire, il n'en est pas ainsi de celle d'identité de genre, qui apporte de la confusion dans le droit. Ne tombons pas dans l'idéologie de la théorie du genre, dans les « iels » et dans tout ce qui vient des États-Unis et qui nous est imposé par une minorité agissante, loin des véritables préoccupations des personnes concernées L'identité de genre d'une personne » est invoquée sans que jamais ce concept ne soit défini. Il est apparu dans des listes de discriminations et s'inscrit dans des lois sans aucune indication sur ce qu'il recouvre. proposition de loi, votée en première lecture à l'Assemblée nationale, ne mentionne pas si la personne concernée est mineure ou majeure. Il s'agit pourtant d'une précision indispensable. Plusieurs spécialistes qui travaillent auprès d'enfants ont alerté sur les dangers d'inclure l'identité de genre dans cette proposition de loi. Cela pourrait empêcher la prise en charge de mineurs souffrant de dysphorie de genre autrement que dans la seule approche transaffirmative. Or, si l'on ne peut nier la détresse de mineurs, en particulier à l'adolescence, qui déclarent ressentir une inadéquation entre leur sexe de naissance et leur sexe ressenti, on ne peut non plus les enfermer dans leur choix en privilégiant une approche transaffirmative prématurée. Aussi, j'ai déposé plusieurs amendements, cosignés par une trentaine de collègues, que je remercie de leur soutien, visant à supprimer la mention d'identité de genre dans cette proposition de loi. Par ailleurs, il m'a semblé essentiel de ne pas oublier d'inclure dans ce texte les thérapies affirmatives de transition sur les mineurs, filles et garçons, qui sont également à interdire. L'un de mes amendements vise donc à punir le fait de prescrire à un mineur, bien

De nombreux témoignages font état des dégâts que causent ces pratiques sur lesquelles nous manquons de recul. À l'heure où des pays très engagés sur le sujet de ce que l'on appelle « la dysphorie de genre » s'interrogent sur leurs pratiques et reviennent à des positions plus prudentes, il est essentiel que la France ne se précipite pas dans la mise en oeuvre de dispositifs qui pourraient porter préjudice aux personnes mineures. La Suède, pays pionnier de la reconnaissance des transgenres, revoit d'ailleurs son protocole vis-à-vis des mineurs. Je tiens également à souligner le danger des réseaux sociaux pour ces mineurs, qui se laissent influencer par les vidéos qu'ils consultent. Cet amendement tend à protéger les mineurs jusqu'à leur majorité. Il est de notre devoir de les préserver. préserver. À l'âge de 18 ans, il sera toujours temps d'engager ce changement de sexe si ces jeunes adultes le souhaitent encore. Non, notre vision de la société n'est ni archaïque ni rétrograde. Elle est réaliste, protectrice et respectueuse.

Nous ne sommes pas non plus en train de légiférer sur les processus de transition des personnes trans, que ces dernières souhaitent avoir recours à des chirurgies, à des traitements hormonaux ou à rien du tout, et cela quel que soit leur âge.

Madame la sénatrice Eustache-Brinio vous souhaitez exclure les personnes trans du champ d'application de ce texte. Dans les faits, pour que tout le monde ait les idées bien claires, cela signifie

pour vous faire devenir une personne que vous n'êtes pas. Si tel était le cas, je puis vous assurer que les personnes trans qui se mobilisent contre vos amendements, tout comme l'entièreté des personnes qui se battent dans ce pays pour la dignité humaine et l'égalité des droits, seraient là pour vous protéger. C'est la grande différence entre nous, me semble-t-il : nos vies ne se ressemblent pas, mais je ne me mobiliserai jamais pour changer la vie des autres, pour porter atteinte à leur dignité ou pour en laisser d'autres continuer à le faire. Personne ici ne demande à personne d'avoir l'empathie nécessaire

les jeunes personnes LGBTQI+ ont trois fois plus de risques de se suicider que les autres. Pourquoi ? Parce qu'on les discrimine, parce qu'on les méprise, parce qu'on leur apprend à se détester, parce qu'on leur dépeint un monde dans lequel ils ne peuvent se projeter. Être soi-même n'est jamais une pathologie ; cela ne se guérit pas. Cela se respecte, cela se célèbre. Les thérapies de conversion ne sont pas des thérapies. Elles ne guérissent rien, parce qu'il n'y a rien à guérir. Elles ne convertissent rien : ce sont des tortures, qui détruisent des vies plutôt que de les accueillir, qui maltraitent des gens plutôt que de les respecter. Ces pratiques doivent disparaître. Voter leur interdiction aujourd'hui est indispensable. C'est un message important que le Sénat doit envoyer non seulement aux victimes, mais aussi à leurs bourreaux. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l'indique l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, les thérapies de conversion en question « se basent sur le postulat que l'homosexualité et la transidentité sont des maladies qu'il conviendrait de guérir

un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) appelait à l'interdiction des « thérapies de conversion », qualifiées, à juste titre, de « pratiques contraires à l'éthique, dénuées de fondement scientifique, inefficaces et, pour certaines d'entre elles, constitutives de torture ». Le Parlement européen a adopté une motion afin de condamner les thérapies de conversion et appelé les États membres de l'Union européenne à légiférer pour les interdire en mars 2018. L'année suivante, la commission des lois de l'Assemblée nationale a constitué une mission d'information sur le sujet. La proposition de loi qui nous est aujourd'hui présentée est issue des conclusions de ce travail, que nous saluons. L'objet principal de ce texte est de créer une infraction autonome relative aux thérapies de conversion. Désormais, le fait de chercher à modifier ou de réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne sera condamné. la création d'un tel délit spécifique est nécessaire pour mieux combattre ces pratiques inhumaines et mieux quantifier les victimes. Mme la rapporteure a redéfini les contours de quelques articles pour simplifier et clarifier l'objet du texte, en précisant, par exemple, que l'infraction n'est pas constituée lorsque les propos répétés de parents ou de professionnels de santé « ont seulement pour objet d'inviter à la prudence et à la réflexion la personne, eu égard notamment à son jeune âge, qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. » Il s'agit là d'un appel à la prudence, qui fait suite à des affaires de poursuites engagées à l'encontre de certains parents bienveillants.

ils ne lui imposent pas d'examiner systématiquement cette question. Or le texte de la commission tend à prévoir que le juge pénal devra se prononcer systématiquement, en cas de condamnation d'un titulaire de l'autorité parentale, sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de cette autorité. craignent qu'une telle disposition n'empêche d'accompagner les personnes qui s'interrogent sur leur identité ou leur sexualité. Au contraire, en définissant les thérapies de conversion dans la loi, nous évitons toute confusion l'article 1 est très précis sur ce qui doit être entendu comme thérapie de conversion. Quant à ceux qui réfutent la notion d'identité de genre et qui refusent de sortir d'une vision binaire et purement biologique du sexe, je me permets de leur rappeler que cette notion est bien définie et installée dans le droit français. Elle a été jugée claire et précise par le Conseil constitutionnel en 2017.

et de souffrances psychiques, parfois physiques. Il est important d'entendre les associations qui travaillent sur ces sujets, d'écouter leur parole et d'entendre l'expression multiple des identités. Pour notre part, nous pensons que, loin de séparer les uns et les autres, de mettre les gens dans des cases bien définies, la reconnaissance de ces identités et leur respect permet de créer du commun dans une société où chacun et chacune peut pleinement s'épanouir. La République et ses valeurs gagneront

comme chacun d'entre nous, en préparant l'examen de cette proposition de loi, j'ai dû lire les témoignages et les récits sidérants de brutalité de ceux qui ont vécu ces prétendues thérapies de conversion. Il est peu de dire que ces actions sont archaïques et fondées sur des idées rétrogrades. Si ces pratiques restent, dans notre pays, largement minoritaires et le plus souvent marginales, elles relèvent toutefois d'un degré de violence morale et physique particulièrement élevé, allant même jusqu'à la torture dans certains cas.

ce qu'il y a de délicat dans cette lutte, c'est que les pratiques peuvent prendre plusieurs formes : thérapies non scientifiques, stages, conférences, entretiens, qui peuvent être accompagnés d'injections de testostérone, de traitements par électrochocs ou encore de diffusions d'images

sont menées sur la base d'idéologies homophobes, pénalement répréhensibles, contraires à la dignité humaine et à la plus intime des libertés individuelles, la liberté sexuelle. la liberté sexuelle. Le groupe RDSE est sensible à cette question depuis longtemps. Le 1 octobre 2019, notre ancienne collègue Françoise Laborde déposait une proposition de loi visant à engager une campagne de prévention et de lutte contre les thérapies de conversion.

Quoi qu'il en soit, je veux dire toute notre satisfaction de voir ce texte inscrit à notre ordre du jour. Il faut saluer la position de notre commission des lois, notamment sur la question du rôle des parents dans l'accompagnement des enfants.

visant à supprimer du champ du dispositif les cas où l'acte aurait lieu en vue de modifier l'identité de genre d'une personne. Je crois que nous ferions une erreur en adoptant une position restreignant le champ de la nouvelle infraction que crée ce texte.

adoptait une résolution exhortant les pays membres de la communauté à interdire les thérapies de conversion censées modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existait en France aucune loi visant à proscrire ce genre de pratiques particulièrement barbares et dont certaines se rapprochent d'actes de torture. Si le phénomène est peu documenté, les rares témoignages connus sont glaçants injections de testostérone, électrochocs et autres psychothérapies forcées composent le quotidien des victimes de ce qu'on appelle communément des « thérapies de conversion Je souhaite m'arrêter un instant sur l'utilisation de ce vocabulaire. Ce terme de « thérapie » induit directement que l'homosexualité serait une maladie, tout comme l'appartenance à un genre sortant du cadre binaire. Cette idée conservatrice est encore prégnante dans une partie de notre société, particulièrement au sein de communautés religieuses extrémistes, qui font de cette doctrine passéiste leur fonds de commerce. Je souhaite adresser un message aux victimes de ces thérapies, ainsi qu'aux personnes tentées de se lancer dans un tel processus : « Vivre libre et en sécurité, c'est votre droit le plus total. Peu importe votre genre ou votre orientation sexuelle. Restez comme vous êtes. Vous n'êtes pas seuls. Les associations sont nombreuses à venir en aide aux jeunes qui éprouvent des difficultés à vivre leur orientation sexuelle ou leur genre. L'État doit maintenant octroyer les moyens nécessaires pour permettre à toutes les personnes LGBTQIA+ de vivre librement. Des accompagnements doivent être proposés dans tous les établissements scolaires, mais aussi hors de leurs murs, aux personnes qui, pour des raisons souvent variées, souffrent de ne pouvoir s'épanouir pleinement du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Ce travail devrait se coupler de campagnes de pédagogie et de sensibilisation aux sexualités et aux droits de toutes les personnes LGBTQIA+

Ce texte était très attendu, et nous nous réjouissons qu'il soit enfin inscrit à l'ordre du jour, après quelques tergiversations du Gouvernement, sur lesquelles je reviendrai.

: si, effectivement, le droit pénal spécial prime sur le droit pénal général, rien n'empêchera demain, après le vote de ce texte, que des infractions voisines des thérapies de conversion soient sanctionnées. Vos craintes en tant que juriste me semblent donc

On le sait, ces pseudo-thérapies produisent des dommages profonds sur la santé physique et mentale des personnes, souvent jeunes, qui les subissent. Elles reposent sur une conception assimilant l'homosexualité et la transidentité à des maladies. Ce n'est pas acceptable,

des thérapies de conversion. En mars 2018, le Parlement européen adoptait une motion condamnant ces pratiques et appelant les États membres à légiférer pour les interdire. Pourtant, en France, bien que l'homosexualité ne soit plus considérée comme une pathologie psychiatrique depuis 1981,

comme véhicule législatif, a ensuite affirmé, lors d'une réponse à une question au Gouvernement en mai dernier, que le droit existant suffisait et qu'une circulaire serait prise. J'ai bien entendu vos propos tout à l'heure et je sais ce que vous avez dit à l'Assemblée nationale. Le contexte a changé, tant mieux.

Comme elles le soulignent, même si le droit pénal permet de sanctionner certaines pratiques, évoquées par notre collègue Philippe Bonnecarrère, telles que l'abus de faiblesse ou les faits de violences, l'arsenal législatif actuel, notamment en raison de son manque de lisibilité, ne suffit pas à lutter contre ces dérives. Non seulement de telles pratiques ont cours sur notre territoire depuis plusieurs années, mais les travaux de la mission d'information de l'Assemblée nationale tendent à montrer leur extension récente et leur caractère protéiforme. qu'un texte réponde à la nécessité de faire évoluer notre droit, en créant une infraction spécifique qui permettra d'identifier clairement ces pratiques et de donner une reconnaissance aux victimes. Je veux saluer le travail très constructif de Mme la rapporteure, qui a utilement complété le texte en prévoyant notamment que, lorsque l'auteur de l'infraction sur un mineur est titulaire de l'autorité parentale, le juge pénal se prononce en cas de condamnation sur le retrait total ou partiel de l'exercice de cette autorité. Si cette possibilité existe déjà aujourd'hui, l'examen systématique va dans le sens d'une meilleure protection des mineurs victimes. Nous approuvons également l'ajout de circonstances aggravantes à l'article 3, afin de punir plus sévèrement les infractions commises par des professionnels de santé à l'encontre d'un mineur ou d'une personne vulnérable. Nous proposerons toutefois des amendements, afin d'améliorer encore cette proposition de loi. Tout d'abord, il nous semble essentiel de veiller à ce que l'accompagnement des personnes en quête de leur identité ne soit pas affecté par ce texte. Aussi, nous souhaitons exclure expressément de son champ les soins et l'accompagnement relatifs au parcours de transition et au changement de sexe. Nous défendrons également la proposition du collectif Rien à guérir d'élargir les préjudices nécessaires pour caractériser l'infraction au fait de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime. La rédaction initiale prévoit l'atteinte à la santé mentale ou physique, préjudice qui peut être parfois difficile à démontrer. Nous considérons que ces pratiques doivent être punies, même lorsque la santé physique ou mentale n'a pas été détériorée. Nous souhaitons également rétablir l'article 2, qui tendait à faire de ces pratiques des circonstances aggravantes aux violences volontaires. Et parce que la proposition de loi passe sous silence le nécessaire aspect de la prévention, nous souhaitons renforcer le contenu des programmes scolaires sur le respect de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Nous sollicitons également un rapport sur les besoins de la médecine scolaire pour accompagner au mieux les élèves victimes de traitements discriminatoires ou de harcèlement, notamment dans le cadre de la vie scolaire. Sur ce sujet, il nous semble important qu'un travail soit mené, afin de pouvoir quantifier, repérer et prévenir. Enfin, il nous semble nécessaire d'associer à ce débat les traitements et interventions visant les enfants intersexes. Il s'agit là, en effet, d'interventions invasives portant atteinte, hors nécessité vitale, aux caractéristiques sexuées de mineurs, actes qui peuvent parfois avoir des conséquences difficiles. Nous espérons que le débat de ce jour permettra de contribuer à faire avancer ce combat pour l'égalité et que nos propositions trouveront ici un accueil favorable. Toutefois, malgré le caractère largement consensuel de ce texte,

De quoi parlons-nous ? De quelque chose qui relève de l'intime et qu'il n'est pas possible de juger. D'une conviction personnelle de se sentir homme ou femme, parfois ni l'un ni l'autre ou les deux à la fois. Ce sentiment peut être en accord avec la réalité biologique ou non. Qui sommes-nous pour juger d'un ressenti, d'une conviction aussi intime ? Je veux ici exprimer la volonté de notre groupe d'affirmer le droit de chacun au cheminement personnel vers son identité. Contrairement à ce que ses détracteurs avancent, la notion d'identité de genre est bel et bien définie. Elle figure déjà dans la loi,

il est aujourd'hui nécessaire de reconnaître ces violences, de reconnaître le statut de victimes à ceux qui les ont subies et, enfin, de permettre qu'elles soient sanctionnées.

le 17 mai 1990, l'Organisation mondiale de la santé marquait un virage aussi tardif qu'historique en supprimant l'homosexualité de la liste des pathologies mentales. Il faudra attendre 1992 pour que la France rejoigne enfin le camp du progrès. Depuis lors, de nombreux progrès ont été réalisés dans notre pays en faveur des droits des personnes homosexuelles. Pourtant, la recrudescence des violences commises contre les personnes LGBT, constatées par SOS homophobie en 2020, témoigne de la persistance d'un sentiment homophobe au sein de notre société. Qu'il s'agisse d'expressions de rejet, d'insultes ou même d'agressions physiques ou sexuelles, ces exactions sont le plus souvent commises dans l'espace privé, à l'abri des regards. Véritables actes de torture, les thérapies de conversion figurent au nombre de ces violences. Qu'elles s'inscrivent dans un contexte médical ou au sein d'un mouvement religieux, qu'il s'agisse de médicaments, d'électrochocs, d'un lavage de cerveau ou même de séances d'exorcisme, les traitements pseudoscientifiques visant à réformer l'orientation sexuelle d'un individu sont toujours traumatisants et suscitent une profonde souffrance chez ceux qui les subissent. C'est pourquoi je salue cette proposition de loi, qui permettra de clarifier définitivement l'interdiction des thérapies de conversion envers les personnes homosexuelles. Certes, ces pratiques barbares pouvaient déjà être poursuivies au titre des violences volontaires, du délit d'abus de faiblesse, du harcèlement moral ou encore de l'exercice illégal de la de la médecine. Mais l'absence d'infraction spécifique rendait difficile le recueil de statistiques judiciaires concernant les thérapies de conversion, donc l'évaluation de l'ampleur du phénomène. De plus, l'autonomisation de la sanction des thérapies de conversion facilitera la prise de conscience des victimes potentielles, en mettant à leur disposition un outil juridique solide sur lequel s'appuyer lors du dépôt de plainte. Enfin, la reconnaissance explicite de l'interdiction des thérapies de conversion permet à la France de s'inscrire en conformité

d'un amendement, par notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio. À l'inverse de la notion d'identité sexuelle, le concept d'identité de genre importé des États-Unis demeure, pour l'heure, une dénomination imprécise, aux contours nébuleux, qui nuit à la clarté du droit. Plusieurs spécialistes ont tiré la sonnette d'alarme quant au risque induit par l'inclusion de la notion d'identité de genre dans la proposition de loi pour les enfants atteints de dysphorie de genre. Ces derniers risqueraient en effet de se retrouver enfermés dans une démarche transaffirmative de façon très prématurée. À cet égard, je conteste le procès en idéologie qui est fait à notre collègue. Bien que la détresse suscitée par la discordance entre le sexe constaté à la naissance et le sexe ressenti ne fasse pas l'ombre d'un doute, il paraît essentiel de ménager le plus longtemps possible la possibilité pour l'enfant de se déterminer sexuellement dans un sens ou dans l'autre. Enfin un peu de

l'État et son personnel politique ne sont pas là pour dire aux Français qui ils peuvent aimer ou non. À vrai dire, nous sommes surtout là pour permettre à chacun de s'épanouir pleinement, et cela en prenant un soin particulier à protéger les plus vulnérables. Cette proposition de loi vise à pénaliser les thérapies dites « de conversion ». En effet, leurs organisateurs, estimant que les personnes homosexuelles sont malades, prétendent pouvoir modifier leur orientation sexuelle. Vous vous en doutez, les premières victimes de ces prétendues thérapies sont très souvent de jeunes adolescents dont les parents n'acceptent pas l'orientation. Oui, il nous faut les protéger, car ils sont vulnérables. Toujours parce que les mineurs sont fragiles, nous devons aussi les protéger de démarches trop hâtives de changement de sexe. En cela, je soutiens les amendements de ma collègue Jacqueline Eustache-Brinio, qui visent à les réserver aux majeurs. Ces démarches sont loin d'être anodines, et nous devons nous assurer qu'elles sont le fruit d'un consentement libre et éclairé du jeune adulte. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de jeter un regard suspicieux sur une telle démarche. Les bloqueurs de puberté et les traitements hormonaux n'ont absolument rien d'anodin, et le chemin inverse est très lourd. L'adolescence est par définition cette période de la vie où l'on se cherche où l'on se perd parfois, mais toujours pour mieux se retrouver. C'est un chemin difficile et je sais qu'il peut être dur à vivre pour certains parents, qui sont témoins de ce mal-être. Mais n'est-ce pas à notre société d'accepter cette période de questionnement plutôt que de vouloir imposer toujours plus vite des choix aussi lourds à de jeunes adolescents ? L'enfer est pavé de bonnes intentions, et nous devons nous garder de tout raisonnement binaire- c'est le cas de le dire. Laissons à ces enfants le temps de se construire, de se choisir, et luttons ardemment contre toutes les formes de harcèlement au sein de nos écoles, car c'est surtout de cela qu'il s'agit. Les amendements de ma collègue Jacqueline Eustache-Brinio visent à supprimer, dans le texte, la notion d'« identité de genre vraie ou supposée J'en suis convaincu, certains militants professionnels penseront qu'il s'agit de rayer cette notion du débat public. Il n'en est rien, et, d'ailleurs, comment le pourrions-nous ? Il est simplement question de préserver notre droit d'une notion confuse Le concept d'identité de genre n'est pas défini. Il est apparu malgré tout dans des listes de discriminations, sans aucune indication sur ce qu'il recouvre, rendant ainsi inopérante l'application des mesures voulues. Il faut comprendre que des notions aussi confuses laissent une interprétation si grande aux juges du fond qu'elles permettent l'arbitraire. Je doute que cela soit l'effet visé Cette proposition de loi, amendée par les amendements que je viens d'évoquer, deviendrait pleinement celle de la tolérance, celle qui refuse que l'on somme une personne de changer son orientation sexuelle, mais aussi celle qui refuse que l'on presse un jeune adolescent de changer de sexe. Je le crois, c'est à notre société d'accepter la différence, les questionnements, les doutes, les interrogations que peut faire naître l'adolescence, et c'est à nous, législateurs, de préserver ce temps si précieux. Je le conçois, certains parents, sûrs de la volonté de leur enfant, trouveront que ce temps offert n'est que souffrance supplémentaire. Mais qu'en serait-il du reste de la vie de cet enfant en cas de changement de sexe précipité ? Cette question doit être posée. Telle est ma position, et c'est à ces conditions que je voterai en faveur de ce texte. La discussion

Une personne transgenre est une personne qui ne s'identifie pas à son sexe de naissance et qui souhaite en changer grâce à un parcours médical et des procédures administratives destinées à modifier son état civil. Au cours de mes auditions, j'ai discuté avec des médecins qui accompagnent des personnes transgenres depuis plus de vingt ans. Des protocoles ont été élaborés, et la Haute Autorité de santé a publié dès 2009 un guide sur la prise en charge du transsexualisme en France.

que les termes « identité de genre » étaient suffisamment clairs et précis pour pouvoir entrer dans le code pénal, sans porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel notait que, en ayant recours à la notion d'identité de genre, le législateur avait entendu viser le genre auquel s'identifie une personne, qu'il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l'état civil ou aux différentes expressions de l'appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin. Compte tenu de cette jurisprudence, l'emploi des termes « identité de genre » dans la proposition de loi ne me semble pas poser de difficulté. Je rappelle d'ailleurs que cette expression figure - là encore, plusieurs de nos collègues l'ont rappelé - dans le code pénal depuis 2016. On la trouve également depuis 2017 dans le code de procédure pénale et dans le code du travail. également inscrite dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le code du sport, dans le code de la sécurité intérieure et dans le code de la santé publique. La proposition de loi ne comporte donc aucune innovation sur le plan sémantique. Dernier élément, Dernier élément, le plus important selon moi : les auditions auxquelles j'ai procédé ont montré que, si l'homosexualité était désormais relativement bien acceptée dans notre société, les personnes transgenres continuent en revanche de se heurter à d'importantes discriminations. Il est donc nécessaire que la loi les protège, et ce serait un mauvais signal que de supprimer les références à l'identité de genre, donc de gommer l'existence de ces personnes transgenres. La commission a cependant été attentive aux préoccupations exprimées par nos collègues, qui craignent que l'interdiction des thérapies de conversion ne rende impossible une approche prudente et mesurée face aux demandes exprimées par certains adolescents. Un parcours médical visant le changement de sexe est éprouvant ; il doit donc être mûrement réfléchi. C'est pourquoi nous avons précisé qu'il n'y aurait évidemment pas d'infraction lorsqu'un professionnel de santé ou un parent, par exemple, invite à la prudence et à la réflexion une personne qui s'interroge sur son identité de genre. Le texte transmis par l'Assemblée nationale était, à mon avis, sans ambiguïté sur ce point, mais nous avons malgré tout voulu ajouter ces dispositions interprétatives pour lever les derniers doutes qui pouvaient subsister.

Elles se sont suicidées parce qu'elles ne supportaient plus le rejet, la discrimination et le harcèlement qu'elles subissaient au quotidien. Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour elles et pour leur famille. Elles étaient toutes des personnes transgenres. Aussi, vous comprendrez que ce gouvernement ne soutienne pas ces amendements, qui ont pour objet de supprimer la notion de genre et de rendre inapplicable le texte aux personnes transgenres, qui sont particulièrement exposées aux thérapies de conversion. Je voudrais vous remercier, madame la rapporteure, de vos explications très riches et très complètes. Je ne reviendrai pas en détail sur la notion d'identité de genre, qui est loin d'être inconnue ou floue, comme je l'ai entendu tout à l'heure. Elle figure déjà dans le code pénal,

Aussi, on ne peut que s'interroger sur l'obstination de la droite sénatoriale à vouloir mener ce que Mme Eustache-Brinio a décrit elle-même comme un combat d'arrière-garde. Pendant longtemps, l'homosexualité a été considérée comme un délit. Il a fallu attendre que la gauche arrive au pouvoir pour que ce délit soit supprimé. nous nous sommes battus pour que le mariage soit ouvert à tous. Aujourd'hui, et c'est une bonne chose, vous avez évolué, puisque vous acceptez l'idée d'interdire les thérapies de conversion. Toutefois, point trop n'en faut

Texte après texte, dans cet hémicycle, depuis un an et demi que j'y siège, j'entends les mêmes utiliser inlassablement la notion d'identité de genre comme un chiffon rouge ou un repoussoir. Mes chers collègues, je voudrais vous dire que cette notion d'identité de genre est documentée depuis au moins les années 1930. Elle a été étudiée par le docteur Magnus Hirschfeld dans le cadre de l'Institut de sexologie qu'il dirigeait et administrait à Berlin. Lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, son institut a été brûlé, et le docteur Magnus Hirschfeld a trouvé refuge ici à Paris, boulevard Arago ; il est mort à Nice, où il est enterré. Ses travaux font autorité depuis au moins les années 1930

Dans la rédaction actuelle sont seulement mentionnés les actes ou paroles « ayant pour effet une altération de [l]a santé physique ou mentale » de la personne concernée. Cela revient, dans les faits, à demander aux victimes d'être capables de prouver une détérioration de leur état. C'est ignorer un élément essentiel dans la qualification des faits par le juge : la volonté de nuire. La volonté de nuire est constitutive de nombreuses infractions, le harcèlement moral

toutes les thérapies de conversion doivent être interdites. C'est pourquoi nous souhaitons ajouter les mots « susceptibles de porter atteinte », afin que la victime n'ait pas de

termes du texte transmis par l'Assemblée nationale, l'infraction est constituée lorsque des pratiques, comportements ou propos répétés visent à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne et ont pour effet une altération de sa santé physique ou mentale. amendements proposent que l'infraction soit constituée si des pratiques, comportements ou propos répétés sont « susceptibles » de porter atteinte aux droits ou à la dignité de la personne et d'altérer son état de santé. L'infraction deviendrait donc beaucoup plus facile à caractériser, mais aussi beaucoup plus large ; il ne serait plus nécessaire de démontrer que la personne a subi un préjudice. Des pratiques seulement « susceptibles » de porter atteinte à la dignité de la personne, ce qui est une notion assez subjective, pourraient être condamnées. me paraît donc raisonnable d'en rester à la rédaction retenue par l'Assemblée nationale : celle-ci garantit que seules des pratiques imposées à la personne et qui nuisent à sa santé physique ou mentale seront sanctionnées et que les accompagnements spirituels que recherchent certaines personnes homosexuelles ou transgenres,

que je viens d'exposer, je crois raisonnable de s'en tenir à la rédaction équilibrée retenue par l'Assemblée nationale : l'infraction est constituée si la victime a subi un préjudice quant à sa santé, mais

Pour les raisons précédemment indiquées, nous avons considéré que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale constituait un bon équilibre. J'ajoute que les comportements, pratiques et propos répétés que l'on rencontre dans le cadre de thérapies de conversion n'ont jamais

l'avis du Gouvernement ? Le principe constitutionnel de légalité impose de définir précisément les éléments constitutifs d'une infraction. J'entends bien sûr parfaitement les objectifs qui sont visés par les auteurs de ces amendements, mais, sur le plan strictement juridique, la notion de « dignité de la personne » n'est pas définie par la loi. J'ajoute que, comme pour tout dommage, il faut pouvoir prouver un préjudice.

euros d'amende. En cas de circonstances aggravantes, les faits visés seraient punis de cinq ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. On pourrait débattre longuement du quantum de peine le plus adapté adapté ; les peines prévues dans le texte qui nous a été transmis par l'Assemblée nationale me semblent déjà dissuasives. Elles sont conformes à ce que la députée Laurence Vanceunebrock avait envisagé dans son texte initial.

Toutefois, les violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime sont sanctionnées d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le quantum des peines applicables au nouveau délit de thérapie de conversion

d'être facteur de confusion, sans améliorer la protection des victimes. Est-il besoin en effet de préciser qu'un parcours de transition visant au changement de sexe ne saurait être assimilé à une thérapie de conversion ? La seule hypothèse qui aurait pu selon nous susciter des interrogations est celle d'un professionnel de santé demandant à la personne qui le consulte d'attendre avant de s'engager dans un parcours de transition, mais il me semble que, en la matière, nous avons levé toute ambiguïté en adoptant, en commission,

les traitements médicaux dispensés dans le cadre d'un parcours de transition. Je le rappelle, l'infraction ne pourra être caractérisée que si les faits ont pour effet une altération de la santé physique ou mentale de la victime. Cette exigence permet de garantir que l'accompagnement des personnes dans le cadre d'un parcours de transition ne pourra être pénalisé sur le

professionnels de santé « ont seulement pour objet d'inviter à la prudence et à la réflexion la personne, eu égard notamment à son jeune âge, qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. En premier lieu, cet alinéa est inutile, dans la mesure où les propos incitant à la réflexion et à la prudence n'entrent pas dans le champ des éléments constitutifs de la nouvelle infraction créée. Les conseils prodigués de manière bienveillante et adaptée ne sont pas susceptibles d'être réprimés, puisqu'il est nécessaire que les propos tenus aient pour effet une altération de la santé physique ou psychique de la victime. En deuxième lieu, cet ajout est vecteur de confusion, dans la mesure où il assimile aux pratiques visant à modifier ou à réprimer l'identité de genre le parcours médical tendant au changement de sexe, lequel n'est pourtant pas concerné par l'infraction créée. En troisième lieu, il n'est pas opportun de créer une cause d'irresponsabilité pénale fondée sur les mobiles de l'auteur, car, en droit pénal,

donc soit superflu soit source d'insécurité juridique. On n'est pas bienveillant quand on cherche à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne ! Si l'on est juste en train d'appeler une personne à la prudence de façon bienveillante

concernant la définition de l'infraction prévue à l'article 1. Nous avons constaté que la création de cette nouvelle infraction suscitait des inquiétudes concernant son impact sur l'accompagnement des personnes transgenres. Des associations craignent, par exemple, que seule une approche consistant à conforter la demande de changement de sexe soit désormais autorisée. Or il arrive que des adolescents s'interrogent sur leur identité de genre sans que leur demande de changement de sexe persiste dans le temps. Il doit rester possible de les inviter à prendre le temps de la réflexion sans que

Enfin, je veux saluer l'initiative de notre rapporteure Dominique Vérien, d'ailleurs suivie par la commission des lois, de rétablir, comme dans le texte initial, la possibilité pour le juge de se prononcer sur le retrait total ou partiel

ou l'identité de genre, vraie ou supposée, de la personne. Il nous semble très important de qualifier ainsi d'éventuelles violences volontaires. Quel est l'avis de la commission ? Le rétablissement ? Le rétablissement des circonstances aggravantes applicables aux infractions, notamment aux violences volontaires commises en vue de modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, ne m'apparaît pas opportun ; c'est d'ailleurs pourquoi nous avions supprimé en effet un facteur de confusion, le juge ayant la possibilité de retenir la qualification de violences aggravées ou d'appliquer la nouvelle infraction autonome créée par l'article 1 de la proposition de loi. Il en résulterait donc un risque de conflit de qualification qui poserait un problème au regard du principe d'égalité devant la loi pénale, les mêmes faits pouvant être punis différemment en fonction des qualifications retenues par le juge. Au contraire, la suppression des circonstances aggravantes consolide la répression des thérapies de conversion autour du nouveau délit autonome, étant rappelé que des poursuites peuvent être engagées pour plusieurs motifs si l'auteur des faits a commis plusieurs infractions.

l'avis du Gouvernement ? Madame la sénatrice, je suis défavorable au rétablissement de cette circonstance aggravante générale, compte tenu des difficultés d'articulation entre celle-ci et l'infraction autonome de l'article 1, qui réprime les thérapies de conversion. conversion. La création d'une telle cause d'aggravation entraînerait des risques de concours de qualification pénale : on ne peut à la fois créer un délit autonome et un délit de violences psychologiques aggravées par l'intention de modifier l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Le Gouvernement a par ailleurs une préférence pour le nouveau délit de l'article 1, qui présente l'avantage d'être beaucoup plus lisible. Il ne peut donc qu'être défavorable au rétablissement de la circonstance aggravante à l'article 2. J'ajoute par ailleurs que le nouveau délit créé à l'article 1 est une porte d'entrée pour le juge,

an. Les parents, accompagnés de médecins, la plupart du temps, doivent déterminer administrativement le sexe de leur enfant, et se déroulent parfois des actes chirurgicaux

vise la question délicate du parcours de transition pour les mineurs transgenres, pour interdire les traitements bloqueurs de puberté, les hormonothérapies et les opérations chirurgicales avant 18 ans. Je suis convaincue comme vous, chère collègue, qu'il faut faire preuve de prudence envers les mineurs qui s'interrogent sur leur identité de genre. Un adolescent peut éprouver un mal-être et l'attribuer à tort à un problème de transidentité. Il faut donc prendre le temps de la réflexion et s'assurer que la demande de l'adolescent persiste dans le temps, avant d'envisager des actes médicaux.

son patient à la réflexion et à la prudence. Je pense toutefois qu'il serait inapproprié d'interdire au détour de cet amendement toute intervention médicale avant l'âge de 18 ans. d'abord, je rappelle que la proposition de loi vise à réprimer les thérapies de conversion, et non à encadrer les parcours de transition. Il s'agit de deux questions bien distinctes, et il serait peu opportun de vouloir modifier les règles encadrant les parcours de transition sans avoir au préalable procédé à un travail approfondi,

aucune audition en ce sens. J'ai simplement entendu un psychiatre et un chirurgien spécialiste des parcours de transition, qui ont souligné à quel point les professionnels de santé étaient précautionneux face à la demande exprimée par un mineur. Le médecin s'assure qu'il est effectivement confronté à un cas de transidentité avant d'envisager un quelconque traitement. Ces spécialistes nous ont également expliqué que les bloqueurs de puberté pouvaient être très utiles. Lorsqu'un adolescent n'est pas à l'aise dans son sexe de naissance, les transformations physiques liées à la puberté peuvent en effet être très mal vécues. Retarder la puberté permet ainsi au jeune à sa famille de réfléchir plus sereinement à la suite de son parcours. Parfois, une hormonothérapie commence, mais ce n'est qu'à partir de 16 ans. Nous devons laisser aux professionnels la liberté d'adapter leur traitement à la réalité de chaque cas. Si des signes de transidentité apparaissent chez un enfant et que le diagnostic est confirmé sans ambiguïté à l'adolescence, pourquoi attendre la majorité avant de commencer un traitement qui va l'aider à mieux vivre ? Je rappelle pour terminer qu'aucune intervention médicale ne peut être décidée sur un mineur

par les médecins et les autres professionnels de santé des personnes en souffrance en raison de questionnements relatifs à leur identité de genre. Elles n'ont rien non plus en commun

Le lien entre ces amendements et la présente proposition de loi n'apparaît donc pas évident. Ensuite, les pratiques que vous évoquez, notamment les traitements hormonaux ou les bloqueurs de puberté, ne visent pas nécessairement le changement de sexe et ne peuvent faire l'objet d'une répression générale, d'autant plus qu'elles font déjà l'objet d'un encadrement légal. La à la bioéthique a ainsi encadré la situation des enfants présentant une variation du développement génital en permettant leur prise en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code de la santé publique.

semble pas inutile ici de faire référence aux enfants intersexes. J'avais d'ailleurs déposé des amendements de même nature sur le projet de loi relatif à la bioéthique.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

rassurer les médecins qui ne feraient qu'accompagner les personnes qui s'interrogent sur leur identité de genre. Nous sommes donc défavorables à ces amendements.